est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 25 octobre 2018 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. J'informe le Sénat que le groupe socialiste et républicain a fait connaître à la présidence le nom de la candidate qu'il propose pour remplacer, en qualité de vice-présidente du Sénat, Mme Marie-Noëlle Lienemann, qui, par lettre en date du 16 octobre dernier, a informé la présidence qu'elle souhaitait démissionner de cette fonction à compter du 1 novembre prochain. La candidature de Mme Hélène Conway-Mouret a été publiée et la désignation aura lieu conformément à l'article 3 du règlement. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la proposition de loi relative à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours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

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, je tiens, en premier lieu, à remercier Catherine Troendlé, auteur de cette proposition de loi, qui a su nous ouvrir les yeux sur une situation qu'il convenait de modifier. Car si les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels sont au coeur de l'action en matière de sécurité civile, ils ne sont pas seuls ! Ils sont accompagnés de plus de 11 000 personnels administratifs, techniques et spécialisés, les « PATS » dans le jargon de la sécurité civile, qui représentent plus de 20 % des effectifs salariés des services départementaux d'incendie et de secours. Ces PATS, fonctionnaires territoriaux pour la très grande majorité d'entre eux, assurent au quotidien l'ensemble des fonctions support nécessaires aux services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS, parfois à un très haut niveau de responsabilité et de technicité. Sans eux, les SDIS ne pourraient pas fonctionner. Certains d'entre eux ont la vie de leurs collègues sapeurs-pompiers entre leurs mains : par exemple, le technicien qui assure le maintien en condition opérationnelle d'un appareil respiratoire isolant est responsable de la sécurité du pompier qui en aura l'usage sur le terrain. Or les PATS ne sont pas représentés au conseil d'administration des SDIS, à l'inverse des sapeurs-pompiers, volontaires ou professionnels. C'est précisément cette injustice que la proposition de loi déposée par Catherine Troendlé vise à réparer. Dans sa rédaction initiale, l'article unique de la proposition de loi tendait à prévoir l'élection par les fonctionnaires territoriaux n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel d'un représentant doté d'une voix consultative au conseil d'administration du SDIS, au même titre que les représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Lors des travaux que j'ai menés pour l'examen de ce texte, cette initiative a été unanimement saluée, tant par les nombreux syndicats qui ont été entendus que par l'ensemble des acteurs institutionnels. Le Gouvernement lui-même a montré son intérêt en engageant la procédure accélérée le 5 octobre dernier. Sur ma proposition, la commission des lois a donc approuvé cette heureuse initiative et a même souhaité aller plus loin dans la reconnaissance des PATS. Ainsi, mes chers collègues, le texte qui vous est soumis aujourd'hui tend à prévoir la représentation des fonctionnaires territoriaux du SDIS qui ne sont pas sapeurs-pompiers professionnels, à l'instar des sapeurs-pompiers, non seulement au conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, mais également au sein de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, la C'est important, car cette commission est consultée sur toutes les questions d'ordre technique et opérationnel- en règle générale, auprès du directeur du SDIS. Le nombre des représentants des PATS au sein de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours serait fixé par voie réglementaire. Il devrait s'élever à deux, comme vous nous l'avez confirmé la semaine dernière Ainsi que le prévoyait déjà la proposition de loi initiale, les PATS disposeraient d'un seul représentant avec voix consultative au conseil d'administration du SDIS, contre deux pour les sapeurs-pompiers professionnels. Comme ceux des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, ce représentant au conseil d'administration du SDIS serait désigné parmi les représentants des personnels administratifs, techniques et spécialisés élus au sein de la commission administrative et technique des services d'incendie et

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureux de revenir devant vous, afin que le Sénat puisse adopter en première lecture la proposition de loi défendue par le rapporteur Loïc Hervé et par la sénatrice Catherine Troendlé,

Ainsi que je le rappelais en commission la semaine dernière, on estime que les services d'incendie et de secours comptaient dans leurs rangs 11 217 personnels des filières administratives, techniques et spécialisées en 2017. Ils représentent près de 22 % des personnels salariés des SDIS. Ces personnels administratifs et techniques, comme M. le rapporteur l'a souligné, ont un rôle essentiel pour le bon fonctionnement des services d'incendie et de secours. Les fonctions support leur reviennent, y compris dans la préparation opérationnelle des interventions des sapeurs-pompiers. En effet, outre les fonctions administratives et financières, ils maintiennent en condition opérationnelle les engins de secours, les matériels de transmission ou encore, M. le rapporteur a cité un exemple, les équipements de sécurité. Comme l'ont souligné les sénateurs qui se sont exprimés en commission, ces personnels ont souvent la vie de leurs collègues sapeurs-pompiers entre les mains. C'est dire si leur rôle est essentiel Cela justifie pleinement que la voix des personnels des filières administratives, techniques ou spécialisées soit entendue au sein des conseils d'administration des services d'incendie et de secours, et que leur représentativité soit encore mieux établie, afin qu'ils soient mieux reconnus. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le cas : ils ne sont pas représentés au sein des conseils d'administration des SDIS. Cette injustice devait être réparée ; je remercie la sénatrice Catherine Troendlé d'avoir travaillé à la rédaction de cette proposition de loi. Les auditions et le travail mené par l'auteur du texte, le rapporteur et les sénateurs de la commission des lois ont permis d'aboutir à la rédaction d'une proposition de loi qui satisfait l'ensemble des groupes. Un amendement déposé en commission par le rapporteur et voté par l'ensemble des sénateurs présents a permis d'intégrer les PATS aux commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours, où ils ont toute leur place également. Le texte ainsi amendé répond aux attentes d'une meilleure intégration des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des différentes instances des services d'incendie et de secours. Ainsi que plusieurs sénateurs l'ont rappelé, le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sur ce texte, afin qu'il soit adopté au plus vite et qu'il entre en vigueur dans les meilleurs délais. Je ne doute pas qu'il sera inscrit rapidement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Je sais que ce texte est également l'occasion pour les sénateurs d'évoquer d'autres préoccupations : vous l'avez largement fait en commission. Je tiens à vous garantir l'implication totale du Gouvernement auprès des sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Nous savons ce qui fait la force du modèle français de sécurité civile, que nous envient tous nos voisins. Nous prendrons une initiative européenne pour préserver le statut des sapeurs-pompiers volontaires dans notre dispositif de secours et leur permettre de concilier leur vie professionnelle et leur engagement citoyen. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, comme cela a été rappelé, cette proposition de loi vise à pallier un manquement concernant les personnels administratifs, techniques et spécialisés, les PATS, qui ne sont pas représentés au sein des conseils d'administration des SDIS. Leur rôle clé et leur nombre justifient que leur voix soit entendue au sein des conseils d'administration des SDIS. Je voterai bien évidemment ce texte. La commission des lois a ajouté une disposition importante, permettant, d'une part, que les personnels administratifs, techniques et spécialisés disposent de représentants à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, d'autre part, que les PATS disposent d'un représentant doté d'une voix consultative au conseil d'administration du SDIS, en qualité de membre élu de la CATSIS, au même titre que les représentants des sapeurs-pompiers. Je salue là le travail de mon collègue rapporteur Loïc Hervé. Je profite de cette intervention pour aborder l'incertitude relative à la transposition de la directive du 4 novembre 2003 dite DETT, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez indiqué à mon collègue Cédric Perrin la semaine dernière que vous alliez proposer dans les prochaines semaines une initiative européenne de nature à garantir que les sapeurs-pompiers volontaires, les SPV, puissent continuer à concilier librement leur engagement et leur activité professionnelle. Vos mots nous rassurent quelque peu. Nous le savons, l'application de la directive impliquerait, notamment, le plafonnement de l'activité cumulée entre travail et volontariat à quarante-huit heures par semaine, l'application du repos de sécurité quotidien entre le travail et l'activité en tant que volontaire, ainsi que le paiement des charges salariales. Autant dire que l'on tuerait le statut de sapeur-pompier volontaire, et donc notre modèle de sécurité civile. Alors qu'ils représentent près de 80 % des effectifs du corps des sapeurs-pompiers, une exemption des SPV du champ d'application de la directive européenne est fondamentale. La revendication au sein de notre hémicycle est forte : la motion de mes collègues Catherine Troendlé et Olivier Cigolotti, adressée au président de la Commission européenne, demandant le rejet de la reconnaissance des volontaires en tant que « travailleurs » au sens de la directive de 2003 dite DETT, a été cosignée par 252 sénateurs. Nous comptons sur votre détermination. Aussi, je tiens à faire remonter une revendication des SDIS concernant les conventions de disponibilité. Les SDIS, et notamment celui de mon département, la Haute-Savoie, soutiennent le développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers à travers ces conventions de disponibilité. Elles permettent à un employeur, public ou privé, de contractualiser avec le SDIS pour une mise à disposition à la carte du salarié, que ce soit pour des interventions, des gardes ou des formations. Cette mise à disposition se fait avec option de subrogation, c'est-à-dire que le SDIS verse à l'employeur le montant des indemnités correspondant au temps de travail non réalisé. Ce dispositif est très performant et assez développé sur notre département, où un label employeur a été mis en place. Il pourrait être judicieux que les employeurs qui contribuent à cet engagement citoyen puissent bénéficier de certains avantages, fiscaux par exemple. Enfin, je soulèverai les difficultés de logement des SPV dans les zones à forte pression immobilière. Ce problème est prégnant en Haute-Savoie. Les jeunes SPV ne parviennent plus à se loger dans les zones très prisées telles que les stations de ski ou la zone transfrontalière. Or c'est justement sur ces bassins que nous avons besoin de maintenir les SPV en astreinte pour couvrir les risques. Les préfectures, conseils départementaux et mairies doivent donc travailler de concert pour trouver des solutions afin de faciliter l'accès au logement local, en contrepartie d'un engagement en qualité de SPV au profit d'un territoire. Je vous remercie pour votre soutien.

nous sommes appelés à légiférer sur une proposition de loi relative à la représentation des PATS au sein des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. chers collègues, comment ne pas s'associer à un texte qui, dans son approche méthodologique- mêlant la procédure accélérée d'initiative gouvernementale à la procédure sénatoriale de législation en commission -comme dans ses nécessaires déclinaisons législatives, met à l'honneur notre Haute Assemblée ? Le groupe La République En Marche, pour sa part, souscrit pleinement aux objectifs assignés par ce texte. Comment ne pas les approuver ? Il importe ici de résorber une rupture d'égalité : alors qu'ils représentent près de 22 % des effectifs salariés des services départementaux d'incendie et de secours et que chacun s'accorde sur le degré d'importance de leurs fonctions institutionnelles, les personnels administratifs, techniques et spécialisés ne disposent pas à ce jour de représentant au sein du conseil d'administration des SDIS, à l'inverse des sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires.

de son rapporteur, Loïc Hervé, la commission des lois a également prévu que les fonctionnaires territoriaux des SDIS qui ne sont pas sapeurs-pompiers professionnels, mais sont très majoritairement des fonctionnaires territoriaux des catégories A, B et C, soient représentés, à l'instar des sapeurs-pompiers et en vertu

L'application de ce principe homothétique dérive directement de la complémentarité fonctionnelle reconnue entre PATS et SDIS, et, comme chacun le sait, de l'importance fondamentale du support administratif dans l'opérationnalité des capacités de projection des SDIS. Les précédents orateurs ont souligné l'importance de leurs fonctions. Le chemin est donc tout tracé ayons l'assurance que cette initiative, à laquelle notre rapporteur a su apporter des gages de crédibilité supplémentaires, ira à son terme. Reste la problématique, soulevée en commission, du principe de répartition des compétences entre l'État et les conseils départementaux l'échelon départemental assure- nous le savons bien ici -le financement budgétaire, en lien avec les communes, d'une politique publique d'obédience étatique et de nature régalienne. Les transferts de charges doivent-ils se traduire, en bout de course, par une participation départementale accrue, non pas financièrement, mais dans le processus décisionnaire ? La réflexion mérite de se poursuivre dans ce domaine, comme dans tant d'autres, où demeurent quelques éléments d'insatisfaction. Cyril Pellevat a évoqué à l'instant, avec le talent qu'on lui connaît, ... Merci ! ... toute la problématique des volontaires.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, cette proposition de loi de bon sens ne peut que recevoir notre approbation, d'autant que les modifications introduites par la commission des lois permettant la représentation des PATS à la commission administrative et technique des SDIS, laquelle débat de questions essentielles d'organisation des services impliquant justement ces personnels

puisque l'occasion m'en est donnée, je rappelle, comme je l'ai fait en commission après Catherine Troendlé, qu'il serait peut-être temps que la concertation, ouverte depuis des années entre le ministère de la santé, en principe responsable des secours sanitaires, et le ministère de l'intérieur, tutelle des

les intervenants juridiquement occasionnels que sont les SDIS sont devenus les principaux acteurs du secours aux personnes, aux frais des collectivités territoriales, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer le peu d'empressement des gouvernements successifs à modifier un aussi intéressant pour lui. Les pompiers refusent d'autant moins de faire le travail que, sur une grande partie du territoire, ils sont les mieux placés et les mieux équipés pour Ce qu'ils demandent, en revanche, soutenus en cela par les élus, c'est d'être au moins correctement défrayés pour le service rendu. Or ce n'est pas le cas, loin de là Non seulement ils sont insuffisamment défrayés, mais ils sont pénalisés lorsqu'ils agissent pour autrui. La promesse faite, par exemple, d'être exonérés du péage des autoroutes n'est toujours pas honorée. Cerise sur le gâteau, les SDIS, comme les autres organismes territoriaux dont le budget est important, devront diminuer leurs dépenses de fonctionnement de 1,2 %. Plus ils feront le travail des autres, plus ils devront faire des économies Je ne sais pas s'ils vont y parvenir ... Quant à la généralisation des plateformes de régulation des interventions sanitaire communes au SAMU, au SDIS et à la police, et autres préconisations que Catherine Troendlé et moi-même formulons depuis quelques années, ... Depuis

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'objet de la présente proposition de loi ne soulève de loi ne soulève aucune difficulté. Les organisations syndicales ont plusieurs fois signalé cette situation incompréhensible que nous allons réparer aujourd'hui. Les personnels administratifs, techniques et spécialisés, les PATS, sont une catégorie professionnelle souvent méconnue, mais qui concourt au service public des sapeurs-pompiers, même s'ils sont cantonnés dans leur bureau ou leur atelier. Ils sont pourtant des membres à part entière de la communauté.

Au même titre que les sapeurs-pompiers, ils montrent un engagement au service de la communauté et de leurs concitoyens. D'ailleurs, il faut le souligner, nombre d'entre eux assurent un service de sapeur-pompier volontaire.

ce texte, fruit d'une réflexion engagée lors des dernières séances de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, et auquel le groupe socialiste et républicain souscrit entièrement. En commission des lois, j'ai défendu, au nom de mon groupe, deux amendements qui ont connu des sorts opposés. Je me réjouis de notre communauté de vues avec le rapporteur au sujet de ce premier amendement. Cela a permis d'étendre l'esprit de ce texte aux commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours. Le second

Nous attendons également une réponse de l'État aux questions soulevées par la directive européenne qui reconnaît les volontaires comme travailleurs. Je salue ici l'interpellation faite par Mme Troendlé et plusieurs de nos collègues sur ce point. Monsieur le secrétaire d'État, pourriez-vous porter à la connaissance du Parlement les conclusions de l'étude des impacts réels pour les services d'incendie et de secours qui est en cours par les services compétents du ministère de l'intérieur, en lien avec le secrétariat général aux affaires européennes ? Il faut protéger l'engagement

? Il ne s'agit pas de nous recroqueviller sur un particularisme local. Nous n'agissons pas par conservatisme. Bien au contraire, protéger la notion d'engagement, c'est promouvoir une valeur qui est consubstantielle à la République.

et de bénéficier de la formation de sapeur-pompier volontaire. Cela a été voté à l'unanimité par la Haute Assemblée. Et cela fonctionne bien ! Préserver notre modèle de volontariat, c'est conforter l'engagement civique, une valeur essentielle pour une citoyenneté active et responsable. Enfin, il faut également lever les freins potentiels à ce don de soi et protéger ceux qui nous protègent. Oui ! À cette fin, je viens de déposer au nom de mon groupe une proposition de loi relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers. Elle vise, selon quelques conditions, à la mise en place d'un anonymat dans le cadre d'une procédure pénale pour inciter les sapeurs-pompiers à déposer plainte lorsqu'ils sont victimes d'agression durant leurs missions. Nous le devons à ces personnes qui nous protègent. Pardon, mes chers collègues, pour la diversité de mes propos, mais tous ces éléments convergent : il faut protéger nos protecteurs Aujourd'hui, nous sommes heureux de soutenir la pierre ajoutée à l'édifice par Mme Catherine Troendlé. Le groupe socialiste et républicain votera donc cette proposition de loi, et continuera à travailler au développement de notre modèle si particulier de secours. La parole est à Mme

service. Eu égard à l'importance de ces personnels, aussi bien en effectifs qu'au regard de leur mission de maintien du matériel qui est centrale, notre groupe a considéré qu'il était indispensable qu'ils puissent être représentés au sein du conseil d'administration des SDIS. SDIS. Dès lors, il nous paraît pertinent que ces personnels soient également présents au sein des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours, puisqu'ils ont à connaître, au quotidien, des enjeux techniques du service. Plus globalement, notre débat doit aussi être l'occasion d'affirmer nos convictions sur l'organisation de nos SDIS. Il nous semble tout d'abord vital et urgent de faire évoluer l'architecture du système de lutte contre les incendies et du secours à la personne dans son ensemble, comme le préconisaient déjà nos collègues Pierre-Yves Collombat et Catherine Troendlé en 2016. Représentante du conseil départemental au sein du SDIS depuis 2015, je fais le même constat depuis plusieurs années, alors que les SDIS sont parfois, malheureusement, le dernier service public dans certaines communes. C'est particulièrement vrai dans le Cantal. Face à la croissance continuelle de leurs charges et à la baisse de leurs recettes, compte tenu du désengagement de l'État et des contraintes budgétaires des départements, les marges de manoeuvre des SDIS se tarissent. Ces derniers ont bien essayé, depuis plusieurs années, d'optimiser leurs moyens, mais cela ne peut suffire ! Le vieillissement démographique et la désertification médicale, avec la fermeture progressive de certains services dans les hôpitaux de proximité, impactent considérablement l'activité des SDIS. Pour illustration, toujours dans le Cantal, le nombre total d'interventions du SDIS a crû de 7 %, tandis que la proportion des secours à la personne a explosé, représentant 79 % des interventions, entre 2016 et 2017. L'appel à l'engagement citoyen de pompiers bénévoles apparaît comme la pierre angulaire d'un système dont le coup d'arrêt pourrait néanmoins bientôt tomber. En France, 79 % des sapeurs-pompiers sont volontaires. Leur présence est au coeur même de notre organisation. Sur les 37 centres de secours du Cantal, les 760 pompiers volontaires permettent d'assurer une bonne partie des interventions dans le département, en complément des 100 pompiers professionnels.

Bien sûr, cette décision est théoriquement circonscrite au cas belge et ne s'applique pas de plein droit en France. Toutefois, nous sommes à la merci d'un recours ... Absolument ! ... devant une juridiction française, qui viendrait totalement remettre en cause notre modèle de secours. Or l'alternative de la professionnalisation à temps partiel du volontariat manque encore de crédibilité, notamment en cas de crise, comme le souligne le rapport de la mission pour la relance du volontariat remis au ministre de l'intérieur le 23 mai 2018. Par conséquent, l'ensemble des membres du groupe du RDSE ont cosigné la motion de nos collègues Catherine Troendlé et Olivier Cigolotti demandant la mise en chantier d'une directive préservant l'engagement volontaire des forces de sécurité et de secours d'urgence.

Vous l'aurez compris, le groupe du RDSE, attentif au bon fonctionnement du service public de lutte contre les incendies et de secours, votera ce texte, dans sa très grande majorité. La parole est à Mme Françoise Gatel, Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi de Mme Catherine Troendlé a donné au Sénat l'occasion d'utiliser une nouvelle fois avec succès la procédure de législation en commission. L'objet du texte s'y prêtait parfaitement. Le groupe Union Centriste affirme son intérêt pour cette procédure moderne et efficace, qui valorise la qualité du travail de commission. N'oublions pas qu'il s'agit là d'une spécificité du Sénat. Elle montre la voie de la modernité et de l'efficacité et pourrait inspirer d'autres assemblées ... Très bien ! La proposition de loi permet de réaffirmer la qualité de nos services départementaux d'incendie et de secours, mobilisés sans relâche, avec dévouement et professionnalisme, pour venir en aide, tout au long de l'année, à nos concitoyens, comme nous l'avons encore vu très récemment, dans des circonstances difficiles. Gardons à l'esprit qu'ils effectuent, en moyenne, une intervention toutes les sept secondes L'examen de ce texte nous donne aussi l'occasion de réaffirmer l'originalité et la très grande valeur du modèle français qui repose sur des sapeurs-pompiers volontaires. Le dernier congrès national des sapeurs-pompiers a d'ailleurs fourni au Gouvernement l'occasion de présenter son plan d'action pour le volontariat, visant à consolider ce modèle altruiste et citoyen et à diversifier le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. C'est une excellente chose. Mais il faudra sans doute aller plus loin pour assurer la pérennité de notre modèle. Tous mes collègues l'ont rappelé : nos sapeurs-pompiers volontaires sont visés, voire menacés par une directive européenne relative au temps de travail, dont l'éventuelle transposition en droit interne pourrait remettre en cause notre modèle de secours français.

Le Président de la République avait d'ailleurs pris l'engagement de « défendre farouchement le modèle reposant sur le volontariat des sapeurs-pompiers qui n'est ni du salariat ni du bénévolat

Certaines de leurs missions sont très techniques. Or de la fiabilité des matériels qu'ils entretiennent dépend parfois directement la vie des sapeurs-pompiers. Leur rôle est donc essentiel. Dès lors, qu'ils puissent être représentés au sein du conseil d'administration paraît légitime. de loi est aussi l'occasion de s'interroger sur l'évolution très importante des SDIS. En effet, le secours à la personne représente aujourd'hui plus de 85 % de l'activité de sapeur-pompier. Cette mission de santé doit être connectée à l'organisation territoriale des soins. La réflexion menée par la ministre des solidarités et de la santé sur la présence médicale dans les territoires ne pourra pas faire abstraction d'une nécessaire articulation entre les services de santé et d'urgence et les missions des SDIS.

Je ne sais si nous devons aller jusque-là. Pour autant, monsieur le secrétaire d'État, nous sommes encore fort éloignés de l'excellent principe du décideur-payeur, et cela pose problème.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en juin dernier, nous avons examiné, dans cet hémicycle, une proposition de loi visant à étendre l'utilisation des caméras mobiles à deux nouvelles catégories d'agents publics, dont les sapeurs-pompiers. Le débat de ce jour concerne la filière administrative et technique des services d'incendie et de secours. Une nouvelle fois, le Parlement se met à l'écoute attentive de ces hommes et de ces femmes qui, au péril de la leur, sauvent, chaque jour, des vies humaines. Il se met aussi au chevet de tous ces sauveteurs, professionnels ou volontaires, personnels administratifs, techniques et spécialisés, qui contribuent à rendre notre société plus sûre, sans toujours en recueillir les lauriers. Rappelons-nous les événements dramatiques de ces derniers mois : ils ont mis ils ont mis en exergue, si besoin était, le rôle éminent des acteurs de la sécurité et du secours, qu'ils soient sapeurs-pompiers professionnels ou qu'ils relèvent de personnels administratifs, techniques et spécialisés. Tous font vivre quotidiennement les mots « mobilisation », « engagement », « entraide », « solidarité Les médias nous rapportent régulièrement le récit d'agressions de pompiers. Oui, du nord au sud et de l'est à l'ouest, nos pompiers sont agressés, caillassés et quelquefois pris à partie par des personnes violentes. En tant qu'élus de la République, nous avons un devoir envers ces personnels. Ce devoir commence par la reconnaissance de tous, y compris des personnels administratifs, techniques et spécialisés, qui représentent un maillon essentiel de la chaîne d'action des soldats du feu. Aujourd'hui, ils sont un élément indispensable des servicesde lutte contre le feu. En 2016, ils étaient 11 200, pour 40 600 sapeurs-pompiers professionnels. Ils occupent des tâches centrales dans la gestion des ressources humaines ou dans le suivi des affaires juridiques. Ils sont aux pompiers ce que les fondations sont à une maison l'élément solide sur lequel repose tout un édifice, toute une institution. Pourtant, ils ne sont pas reconnus. Au sein des services départements d'incendie et de secours, ils n'ont pas voix au chapitre, alors que les sapeurs-pompiers, volontaires comme professionnels, disposent de deux représentants, avec voix consultative. Le dialogue social doit prendre une nouvelle dimension au sein des commissions administratives et des conseils d'administration des SDIS, permettant de lever les éventuelles incompréhensions et de prévenir les conflits.

Au sein des instances de ces services départementaux et des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours, ils pourront alors faire entendre la voix de ces milliers d'hommes et de femmes ayant des missions

les préfets la nécessité d'appliquer les dispositifs de convention opérationnelle existants, qui visent à renforcer l'échange d'informations, à permettre des interventions conjointes avec les forces de l'ordre dans les secteurs les plus sensibles et à faciliter le dépôt de plainte en cas d'agressions. Cet élément est extrêmement important.

Si l'épisode de grande sécheresse qui sévit sur notre territoire depuis le printemps dernier commence tout juste à se clore, nous savons en revanche que ses conséquences risquent, hélas, de fragiliser encore nos agriculteurs dans les mois qui viennent. En effet, cet événement climatique a été d'une telle ampleur qu'il a rapidement plongé de nombreuses exploitations dans la difficulté, avec, en particulier, un effet domino pour les producteurs de fromages. Dans le Cantal, la sécheresse a eu pour premier effet d'obliger les éleveurs à acheter prématurément du foin, dont le coût pèse très lourdement sur les trésoreries. Malgré cette charge, la plupart des exploitants se sont approvisionnés en fourrages pour faire face à leurs besoins. Néanmoins, beaucoup d'entre eux doivent maintenant renoncer à leur niveau habituel de production de fromages, faute d'un bon pâturage au cours de l'été. Je pense au Salers, notamment, dont le cahier des charges impose une herbe de qualité pour la nourriture des vaches. Monsieur le ministre, je salue les annonces que vous avez faites la semaine dernière ici, au Sénat, sur les aides nationales qui viendront en complément des dispositifs européens destinés à alléger les charges des exploitants. Nos exploitants ont vraiment besoin d'un soutien rapide et efficace. Je souhaitais toutefois vous interroger sur ce qui pourrait être fait en amont pour limiter les effets de ces sécheresses, qui, on le sait, risquent d'être récurrentes en raison du réchauffement climatique.

je voudrais tout d'abord vous remercier pour le travail que vous effectuez au sein de la Haute Assemblée sur ces sujets. Je me suis déjà exprimé la semaine dernière. Comme je l'avais dit, l'État est au rendez-vous de la sécheresse que subissent les agriculteurs. Des mesures ont été annoncées, notamment l'exonération

qui est aujourd'hui majeur pour notre agriculture. Le réchauffement climatique et la dérégulation du climat sont là ; il nous faut donc nous soucier de la ressource en eau. Vous avez eu raison, madame la sénatrice, de

le Sénat ce matin. Monsieur le Premier ministre, vous venez de présenter un vaste plan de destruction de la fonction publique par la baisse des effectifs et la fragilisation du statut. Ce plan poursuit le vieux rêve d'un État faible face au jeu des intérêts privés. Que proposez-vous ? Cinquante mille fonctionnaires d'État en moins, après une baisse de 11 % depuis vingt ans, une casse du statut avec un appel massif aux contractuels. la France ne peut se gérer comme une start-up, les règles du service public et le sens de l'intérêt général ne sont pas compatibles avec l'objectif de rentabilité. Votre plan impose aussi une réduction de 70 000 postes dans la fonction publique territoriale. C'est un non-sens : chacun sait que la défaillance du service public d'État est prise en charge par les collectivités locales. D'ailleurs, les points de contact que vous annoncez existent déjà, ce sont les mairies Monsieur le Premier ministre, votre plan libéral est en totale contradiction avec les besoins de notre société. Quand admettrez-vous que la casse du service public, de ce qui ne se marchandise pas, brise le trait d'union, la solidarité sociale territoriale au sein de notre République ? Monsieur le Premier ministre, la voie que vous avez choisie est sans issue, et elle interroge sur l'avenir de notre pays et de l'Europe. Nous attendons de votre part un sursaut républicain pour stopper la saignée que vous imposez aux services publics nationaux et locaux. Allez-vous y mettre fin ?

privé. Nous accompagnerons ces transformations d'une réorganisation du réseau territorial. Le Premier ministre nous a donné une consigne : privilégier l'échelon départemental comme moyen d'action. Vous le savez, à la suite d'interventions de nombreux élus de la Loire, nous avons notamment pris la décision

y regarde de plus près, elles sont bien loin de servir à mettre en place une fiscalité écologique ; il y a même des désengagements dans ce domaine. Elles servent plutôt à boucher les trous des cadeaux fiscaux donnés, dans la première année du quinquennat, aux plus riches. La fiscalité que vous déployez est injuste, elle est punitive. Ces taxes frappent indistinctement les plus fragiles.

avez-vous mis à l'étude une TICPE flottante, comme cela s'est fait il y a quelques années ?

Monsieur le ministre d'État, ce n'est pas parce que l'on peint un matraquage fiscal en vert qu'il devient écologiste ! Car c'est un matraquage fiscal !

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur. Samedi 27 octobre, à Pittsburgh, un terroriste est entré dans la synagogue Tree of Life et a vidé les chargeurs de sa kalachnikov en criant : « Tous les juifs doivent mourir », perpétrant le pire attentat antisémite de l'histoire américaine. Deux jours plus tard, à Paris, une élève de médecine portait plainte contre un certain nombre de ses camarades qui, au nom d'un humour répugnant, voulaient baptiser leur week-end d'intégration « Auschwitz 2019 » ou encore « Rafle 2019 ». Ils illustraient leur proposition d'une photo d'un étudiant juif brûlant dans les flammes. Rappelons-nous aussi les meurtres ignobles de Mireille Knoll et Sarah Halimi, l'attaque sanglante de l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes, l'insoutenable tuerie de l'école Ozar Hatorah à Toulouse, l'assassinat atroce d'Ilan Halimi en banlieue parisienne. Tous furent assassinés parce qu'ils portaient dans leur coeur l'étoile de David. Les mots nous manquent pour répondre à la haine meurtrière qui se déverse sur le sol de la République et fait trembler les remparts de la démocratie. Il est pourtant de notre devoir de prendre la parole et d'alerter la société tout entière contre la recrudescence d'un antisémitisme sanguinaire, dont la Shoah, ignominie de l'histoire de l'Humanité, reste le plus terrible témoignage. Depuis plus de dix ans, une nouvelle vague d'antisémitisme sévit en France, et la France, trop souvent, reste impuissante. Les marches blanches ne suffisent plus, les manifestes restent sans portée, le devoir de mémoire s'essouffle ... Monsieur le ministre, quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre pour combattre l'antisémitisme rampant qui sème la honte, le deuil et l'horreur au pays des droits de l'homme ?

aux proches des victimes, à ceux qui sont meurtris par ces attaques insupportables. Personne ici, personne, n'oublie les attentats, les violences et les insultes dont le seul motif était l'antisémitisme. Personne ici n'oublie les attaques que vous avez évoquées. Personne ici n'oublie le gang des barbares, si bien nommé, qui a assassiné et torturé Ilan Halimi. Pour reprendre les propos du Président de la République,

Nous savons tous que, trop souvent, les victimes ne veulent pas forcément porter plainte, alors même que l'objectif du combat contre l'antisémitisme passe par une condamnation forte, rapide, puissante. Nous avons donc décidé, et c'est une première réponse, de mettre en place le dépôt des préplaintes en ligne pour les infractions discriminantes

total du Gouvernement, des services de l'État, des services de police et des services de la gendarmerie pour lutter contre l'antisémitisme. Si, pour citer Hannah Arendt, « De tous les maux qui ont ravagé le XXsiècle, l'antisémitisme est le seul qui, au fond, demeure incurable », notre combat permanent contre ce mal permettra de le faire reculer.

Monsieur le ministre, vous le savez mieux que quiconque, dans une Europe et un monde pleins de tensions, la diplomatie est l'art de jeter des ponts qui permettent le dialogue au-delà des différences. Voilà qui devrait conduire à bannir toute forme de propos inutilement blessants pour nos interlocuteurs dont la légitimité démocratique n'est pas contestable, même si le résultat ne nous plaît pas. Malheureusement, quand j'écoute certaines déclarations du Président de la République, je doute de notre capacité à être ceux qui maintiennent le lien et qui unissent. C'est pourtant le rôle que la France a toujours assigné à sa diplomatie. Est-il constructif de déclarer à propos de deux dirigeants européens : « Ils ont raison de me voir comme leur principal opposant » ? Est-ce le rôle du chef de l'État de parler de certains de ses collègues européens en ces termes : « Que font ces esprits fous » Un Président ne devrait pas dire ça ! Le combat contre le nationalisme est un vrai combat. C'est un combat exigeant. Il s'agit de mettre toutes nos forces dans la reconstruction d'une Europe exigeante sur les valeurs, qui doit à la fois panser les plaies d'un divorce douloureux, écouter les peuples et se consacrer aux grands projets. Depuis quelques mois, nos relations avec nos voisins européens se sont dégradées. Au-delà de l'Europe, les tensions demeurent avec la Russie, et après un départ en fanfare aux côtés de Donald Trump, la réalité aujourd'hui est bien différente. Monsieur le ministre, vous êtes connu pour votre sens de la mesure et pour votre habileté. Le Breton que vous êtes sait qu'il faut contrôler ses émotions si l'on veut être respecté et efficace. Ne croyez-vous pas que la voix de la France a beaucoup à perdre si elle se laisse trop souvent aller à l'anathème de la bouche même de son Président ?

Le premier était celui du Président Trump, qui a expliqué comment il fallait progressivement détruire l'ensemble des éléments du multilatéralisme et comment le rapport de force bilatérale devait régenter les relations internationales.

Ce discours a été très applaudi par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement présents. Non, madame la présidente, la diplomatie française n'est pas isolée.

du Président de la République que se tiendra le forum de la Paix, lequel réunira dans quelques jours à Paris plus de 70 chefs d'État et de gouvernement pour reconstruire la paix ensemble. C'est enfin sur l'initiative du Président de la République que se sont tenues les conférences et les

Monsieur le ministre, les discours sont l'apanage du Président de la République. Il est très fort pour faire des discours et pour recueillir l'approbation des auditoires auxquels il les délivre. Mais où sont les actes ?

ma question, à laquelle j'associe notre collègue Nathalie Goulet, à qui ce sujet tient à coeur, s'adresse à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Le 20 octobre dernier, Qader Daoudzai a été tué dans une attaque suicide à Kaboul. suicide à Kaboul. C'était un ancien interprète de l'armée, du temps de sa présence en Afghanistan. La victime s'apprêtait à demander un visa pour la France, après un premier refus en 2015. En effet, lui et toute sa famille étaient menacés de mort par les talibans du fait de son travail pour la France. Il ne pouvait ni retourner dans son village ni sortir de Kaboul. Ses proches ont rapporté qu'il répétait souvent : « Si je ne vais pas en France, je vais mourir dans une attaque ou quelqu'un me tuera ». En 2015, il avait fait état de ces menaces dans sa demande de visa pour la France, qui lui avait été refusée, comme ce fut aussi le cas pour 151 autres personnes faisant partie des personnels civils de recrutement local. Avant sa mort, Qader préparait son dossier pour une nouvelle demande de visa dans le cadre de la procédure dite de « relocalisation » récemment ouverte. Aujourd'hui, ses enfants âgés de deux, trois et quatre ans, désormais orphelins, se trouvent dans un pays en guerre. Plus de 600 auxiliaires de nos forces armées dans le monde risquent ainsi leur vie pour la France. En Afghanistan, ils étaient les intermédiaires indispensables des militaires français auprès des populations. Avant de quitter le pays, la France s'était engagée à les protéger. Elle avait promis de ne pas les oublier. Or force est de constater que la France les a, à l'évidence, oubliés. Il a fallu un mort de plus pour que nous les fassions sortir de cet oubli. Monsieur le ministre, je vous poserai donc deux questions très simples. Quand allez-vous enfin accueillir la famille de Qader Daoudzai ? Que comptez-vous faire pour protéger les auxiliaires locaux de nos armées ?

Ces mesures ont suscité de grandes espérances au sein de la population réunionnaise et auprès des élus réunionnais, tous unis autour de cet enjeu essentiel pour La Réunion.

Deuxièmement, elle a précisé qu'un dispositif au moins équivalent- j'insiste sur les termes « au moins équivalent » financera, à partir de 2020, l'accession sociale à la propriété et la rénovation des logements des propriétaires occupants sous condition de ressources. est venue à La Réunion la semaine dernière. Elle a pu constater à quel point la question du logement est essentielle et nécessite des solutions innovantes et concrètes. C'est pourquoi je la félicite tout particulièrement d'avoir intégré la rénovation dans cette mesure.

Ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé. Depuis quelques jours, la pénurie de médicaments et de vaccins fait la une des journaux. Des associations de malades de Parkinson ont en effet lancé un cri d'alerte, le 28 octobre dernier, pour dénoncer les ruptures de stock qui se multiplient et réclamer un « plan d'action urgent Malheureusement, le problème n'est ni nouveau ni circonscrit aux traitements contre la maladie de Parkinson. En 2017, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a reçu 530 signalements de rupture de stock ou de difficulté d'approvisionnement pour des traitements dits « essentiels », comme les anticancéreux. En dix ans, ce chiffre a été multiplié par dix. Les difficultés touchent aussi bien les médicaments d'intérêt majeur que ceux d'usage quotidien ou les vaccins. J'ai pu discuter directement avec un pharmacien de mon département, qui dépeint une situation difficile. Il est souvent contraint de recourir à des traitements alternatifs pour répondre aux besoins urgents des patients. Un rapport du Sénat, publié le 27 septembre dernier, a mis en lumière l'ampleur du phénomène ; trente propositions Parmi les premières causes de ces ruptures de stock se trouvent les difficultés d'approvisionnement en matières premières, liées à la perte d'indépendance sanitaire française et européenne : 40 % des médicaments commercialisés dans l'Union européenne proviennent de pays tiers et, surtout, 80 % des fabricants de matières premières sont situés en dehors de l'Union. Ces chaînes Ces chaînes de production sont fragiles, notamment dans un contexte de demande exponentielle en technologie de haut niveau. La production française, de son côté, fait face à des difficultés majeures liées à la baisse des prix et à la lenteur du processus d'autorisation de mise sur le marché. La gestion des pénuries déstabilise l'organisation des soins et génère des coûts financiers élevés. Elle met également en danger la santé des patients et leur confiance dans notre système de santé. Aussi, compte tenu de l'expertise de pointe de la France en matière d'innovation médicale et pharmaceutique, pouvez-vous me dire quelles mesures envisage le Gouvernement pour recouvrer une indépendance et une stabilité dans la chaîne du médicament en France et en Europe ?

Les causes des ruptures de stock de médicaments, ainsi que les tensions d'approvisionnement, ont des origines multifactorielles susceptibles d'intervenir tout au long de la chaîne de production et de distribution. le Sinemet, il s'agit de la fermeture du site de production de produits finis aux États-Unis pour une mise en conformité à la fois du produit et du site. Pour faire face à ce phénomène, la France a mis en place un arsenal juridique et a engagé des actions, y compris à l'échelon européen. Depuis 2016, un cadre juridique a été élaboré pour lutter contre les ruptures d'approvisionnement à l'échelle nationale et garantir l'accès de tous les patients à leur traitement, grâce à la mise en oeuvre de nouvelles obligations incombant aux acteurs du circuit de fabrication et de distribution. Néanmoins, et vous avez raison de le souligner, on ne peut se satisfaire de la situation actuelle. Il faut avancer vers la mise en place d'un plan d'action pour lutter contre ces ruptures. Nous souhaitons nous appuyer sur le rapport sénatorial issu des travaux de la mission d'information sur la pénurie de médicaments et de vaccins, publié le 2 octobre dernier Il faut notamment agir sur trois axes : renforcer la coordination nationale et la coopération européenne ; rétablir la confiance entre tous les acteurs de la chaîne pharmaceutique et les usagers par des mesures de transparence et d'information ; enfin, travailler avec les autres ministères et les industriels pour avancer sur la question du désengagement

Je roule au diesel tant que je peux payer le plein- voilà trois ans, on nous encourageait à acheter un véhicule diesel ... Je fume des Gauloises. Je me chauffe au fioul tant que je peux payer le remplissage de ma cuve. Je ne peux plus me faire soigner.

Difficile de croire qu'il s'agirait d'un chômage volontaire, contrairement à ce que l'on peut parfois entendre. On trouve de la souffrance et des ruptures de vie

pays européens, la France est vingt-quatrième pour le taux de chômage. Monsieur le Premier ministre, les chiffres sont têtus et le Président de la République, après dix-huit mois de mandat, ne saurait camper sur une politique qui ne porte pas ses fruits. Pour s'attaquer au chômage, il faut retrouver notre compétitivité économique. La dépense publique est trop élevée dans notre pays. Or, dans la lignée de votre prédécesseur, vous continuez de la faire croître. pourtant bien cette dépense publique hors norme qui plombe durablement notre capacité à revenir au plein-emploi. La hauteur de la dépense publique n'obéit à aucune loi universelle et intangible. Elle indique un choix de société, donc un choix politique.

le chômage de longue durée est un problème auquel le Gouvernement apporte une attention toute particulière. Je veux d'abord rappeler quelques chiffres : depuis plus d'un an,

et ne proposent pas d'offres d'emploi, ce qui alimente ces spirales. Il ne faut pas se tromper, ce problème est d'ordre structurel : même lorsque la croissance repart et que les entreprises cherchent à recruter, une part significative de nos concitoyens ne parvient pas à retrouver un emploi. À ce problème structurel, nous apportons une réponse structurelle, basée sur les compétences et la qualification. Le plan d'investissement dans les compétences va ainsi permettre de former 1 million de chômeurs non qualifiés d'ici à la fin du quinquennat, dont beaucoup sont enfermés dans le chômage de longue durée depuis longtemps. Lutter contre le chômage de longue durée, c'est aussi apporter des réponses innovantes aux personnes les plus en difficulté, notamment les bénéficiaires du RSA. Pour cette raison, dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, nous allons mettre en oeuvre une garantie d'activité qui permettra d'apporter des réponses adaptées aux situations de chacun. D'ici à la fin du quinquennat, 100 000 personnes bénéficieront des aides au titre de l'insertion par l'activité économique. Enfin, ces réponses passeront également par l'appel à projets 100 % inclusion que nous avons lancé et dont les premiers lauréats seront dévoilés dans quelques jours. Là aussi, l'enjeu consiste à trouver des solutions qui prennent en compte la diversité des personnes et des parcours en faisant confiance aux acteurs et aux territoires. Parce que personne n'est inemployable, nous faisons le pari de l'investissement social.

Ma question s'adressait à Mme la ministre du travail. Avec une baisse de crédits de plus de 2 milliards d'euros, le ministère du travail est le grand perdant du budget pour La formation professionnelle semble être la première victime de ce désengagement de l'État. Faute de moyens et de soutien suffisants, l'AFPA- l'Association nationale

ne subventionne pas l'emploi, mais investit dans les compétences et l'insertion des plus vulnérables ». Curieuse manière d'investir dans les compétences lorsque l'on décide de sacrifier le plus gros organisme de formation français Malgré quelques points à améliorer, un récent audit en a souligné les nombreux atouts : un service ouvert à tous, une prise en charge individualisée, un savoir-faire élevé en matière d'ingénierie de formation et un fort taux de retour à l'emploi, en particulier dans l'industrie et le BTP. En 2016, le gouvernement précédent avait voulu ancrer cette structure dans le service public de l'emploi en la transformant en Agence nationale pour la formation professionnelle, professionnelle, avec un statut d'EPIC. Aujourd'hui, force est de constater que l'actuel gouvernement ne semble pas vouloir poursuivre dans cette voie. Quelle est la cohérence entre les paroles et les actes lorsque le Gouvernement prétend vouloir faire de la lutte contre le chômage sa priorité et décide, dans le même temps, de démanteler le service public de la formation professionnelle ?

Ne vous en déplaise, il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver un emploi : il faut être bien formé et bien accompagné. C'est justement ce que fait l'AFPA et ce qui est mis en péril aujourd'hui.

Pour autant, la santé de tous nos compatriotes est aujourd'hui singulièrement mise en danger. En effet, vous ne pouvez ignorer que les cas de contamination par la bactérie sont en constante augmentation. Ces contaminations sont principalement induites par certaines pratiques d'abattage rituel lors desquelles l'animal, dont la gorge est tranchée sans étourdissement préalable, régurgite son contenu stomacal et, dans un instinct de survie, le réingère puis le régurgite de nouveau. Il y avait longtemps ! Bien évidemment, le poste d'abattage ainsi totalement souillé n'est pas désinfecté après chaque opération. Je souligne que les individus les plus fragiles- enfants et personnes âgées -sont les principales victimes d'. Cette affection Cette affection se traduit au mieux par des vomissements et des diarrhées sanglantes, au pire dégénère en un syndrome hémolytique et urinaire pouvant conduire au décès de la personne atteinte. Cependant, malgré les risques avérés, les consommateurs sont tenus dans l'ignorance du mode d'abattage de l'animal dont ils se proposent d'acquérir une pièce de viande. Je ne puis omettre dans mon propos d'évoquer également les risques encourus par tous les maires du territoire s'il advenait qu'une cantine scolaire dont ils ont la charge serve un produit carné infecté. Leur responsabilité pénale serait alors dramatiquement engagée. Aujourd'hui, quiconque achète de la viande court le risque de mettre sa santé gravement en danger, les pouvoirs publics se refusant toujours à délivrer une information pourtant légitime. Dans cet unique souci de transparence et de sécurité pour les consommateurs, le Gouvernement envisage-t-il de rendre enfin obligatoire l'indication du mode d'abattage, afin que nos compatriotes disposent de l'information nécessaire lors de leurs achats ? La parole

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur du débat disposera d'un temps de parole de huit minutes

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la question migratoire est aujourd'hui au coeur des difficultés que traverse l'Europe.

L'afflux des réfugiés vers l'Europe a des causes bien connues : la pauvreté et l'absence d'espérance d'une vie décente en sont l'une des raisons. Mais les crises politiques et les persécutions infligées par des régimes dictatoriaux ont, hélas, aggravé ce phénomène. en Syrie, pays martyr aux 400 000 morts et aux 6 millions de réfugiés, a poussé des centaines de milliers de personnes hors de chez elles. Samedi dernier, j'étais, avec un certain nombre de mes collègues, au Sud-Liban, dans le camp d'Azzieh, auprès de réfugiés syriens de la région d'Idlib. Ces familles ont tout perdu : leur maison, leur terre, leurs proches. Elles survivent grâce à la générosité du Liban, grâce au Haut-Commissariat pour les réfugiés. Elles ne veulent qu'une seule chose : rentrer chez elles. Mais comment imaginer un tel retour aujourd'hui ? La guerre en Syrie est à la croisée des chemins. Souhaitons que le dernier sommet d'Istanbul concrétise enfin un premier pas vers la paix. Dans le même temps, le chaos en Libye a permis à des filières de migration massive de s'installer en Méditerranée, pour faire du trafic d'êtres humains, mêlant réfugiés et migrants, broyant des milliers de vies dans la misère. L'ampleur de cette crise migratoire a remis en cause les principes européens les plus essentiels, comme la solidarité entre États membres ou la liberté de circulation au sein de l'espace Schengen. Depuis trois ans, l'Union européenne a réagi en renforçant les moyens d'action de FRONTEX et les contrôles aux frontières extérieures. La coopération avec les pays tiers, illustrée par l'accord passé en 2016 avec la Turquie, et développée, depuis le sommet de La Valette, avec les pays africains et du pourtour méditerranéen, a progressé. Toutefois, les résultats sont inégaux. Ces mesures ont certes porté leurs fruits : les arrivées en Europe par la Méditerranée sont passées de plus d'un million en 2015 à 172 000 en 2017. Les flux ont diminué de 40 % par rapport à 2017. N'allons pas croire pour autant que le problème des migrations est derrière nous. Il n'en est rien, c'est même tout le contraire. Tout d'abord, on le sait, les passeurs trouvent de nouvelles routes. Depuis la relative fermeture de la voie libyenne, on constate une reprise des traversées entre le Maroc et l'Espagne, alors que cette route dite « de Méditerranée occidentale » était délaissée depuis plusieurs années. Ce flux, endigué par l'action résolue des autorités marocaines, aujourd'hui en première ligne, représente désormais la moitié des traversées vers l'Union européenne. En outre, on constate aussi une augmentation des traversées en Méditerranée orientale, où nous sommes tributaires de la bonne volonté des autorités turques. Car l'Europe, espace de paix et de prospérité, reste une destination de prédilection pour de nombreux candidats à l'émigration économique, particulièrement en Afrique de l'Ouest ou au Sahel. Dans ce contexte, monsieur le ministre, l'Union européenne doit agir ! Pour agir à la source, nous devons aider les pays d'origine et de transit à mieux contrôler la gestion de leurs frontières et à lutter efficacement contre les trafiquants. L'exemple réussi du Niger illustre les résultats qu'il est possible d'obtenir. Ce pays consacre 20 % de ses dépenses budgétaires à la sécurité. La France et l'Union européenne ont raison de le soutenir ! En revanche, j'avoue mon scepticisme s'agissant des plateformes de débarquement mises en avant lors du Conseil européen de juin dernier.

Enfin, l'accent doit être mis sur l'amélioration de nos politiques en matière de renvoi des migrants déboutés en situation irrégulière. Comment se satisfaire d'un taux d'exécution des mesures d'éloignement de 36 % à l'échelle européenne et de 14 % seulement au plan national ? S'attaquer sérieusement à ce problème, c'est envoyer un message de fermeté et asseoir la crédibilité de notre politique migratoire. Nous avons des leviers. Je pense en particulier aux visas. Ayons le courage d'un dialogue ferme et exigeant avec les pays sources, qui ont, eux aussi, besoin de garder leur jeunesse, laquelle constitue leur avenir. Monsieur le ministre, sur ces sujets essentiels, nos concitoyens attendent des réponses fermes, à la fois du Gouvernement français et de l'Union européenne. De grâce, ne les décevons pas ! La parole

auteur de la demande. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les flux migratoires vers l'Europe sont sensiblement moins importants qu'il y a trois ans, même si la vigilance s'impose sur la route de la Méditerranée occidentale, les arrivées en mer par l'Espagne ayant nettement augmenté au cours des derniers mois. Pour autant, jamais les États membres n'ont paru aussi divisés sur la façon d'y faire face. Les États les plus solides sont eux-mêmes confrontés à des tensions politiques internes, on le voit en Allemagne. La crise migratoire, latente, qui avait déjà failli emporter Schengen à la fin de l'année

Depuis le pic de la crise, nous avons indéniablement progressé, mais l'Union européenne a trop souvent réagi dans l'urgence. Une vision d'ensemble lui a manqué. Le Conseil européen du 28 juin dernier, pour surmonter les divisions européennes, s'est entendu sur deux concepts des « plateformes régionales de débarquement » et celui des « centres contrôlés », envisagés comme des instruments complémentaires de la solidarité européenne, à la fois entre les États membres et à l'égard des migrants. L'indispensable respect du droit international dans leur mise en place ne saurait s'affranchir d'une distinction entre les réfugiés et les migrants motivés par des considérations économiques. Ces derniers se trouvent généralement en situation irrégulière. Ils doivent donc être reconduits dans leur pays. Telle est la position que la commission des affaires européennes a exprimée récemment, en adoptant une proposition de résolution européenne sur les réformes de l'espace Schengen qu'il convient de poursuivre. Les conclusions du Conseil européen du 18 octobre dernier ne faisant mention ni des plateformes de débarquement ni des centres contrôlés, je m'interroge, monsieur le ministre, sur le devenir

des travaux de la Commission européenne, laquelle, dans le cadre de ses dernières propositions, cherche à établir un lien entre le renforcement du contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne, notamment FRONTEX, et les politiques d'asile, d'immigration et d'intégration. Ces questions doivent faire l'objet d'une approche intégrée. À cet égard, je me réjouis de l'annonce de la création d'une conjointe auprès du Centre européen pour la lutte contre le trafic de migrants mise en place au sein d'Europol. Les activités de cette agence font du reste l'objet d'un contrôle politique, auquel notre commission contribue activement au sein du groupe de contrôle parlementaire conjoint. Nous y sommes en effet représentés par nos collègues Jacques Bigot l'Union européenne ne réussira pas à répondre durablement à la crise migratoire sans contribuer de façon plus ambitieuse au développement du continent africain.

telle réponse, qui vise forcément le long terme, doit être amplifiée. À cet égard, quels sont, monsieur le ministre, les objectifs que l'on peut raisonnablement fixer au sommet prévu entre l'Union européenne et la Ligue arabe, qui sera organisé par l'Égypte en février prochain ? La parole est à M. le ministre.

Monsieur le président, monsieur le président Cambon, monsieur le président Bizet, mesdames, messieurs les sénateurs,

et des préoccupations que nous partageons avec nos partenaires européens. En 2015, 1,8 million de personnes avaient franchi de manière irrégulière les frontières extérieures de l'Union. Depuis lors, la situation a considérablement évolué, les franchissements irréguliers ayant fortement décru. Les initiatives prises à l'échelon européen ont donc porté leurs fruits, puisque, entre le 1 janvier et le 21 octobre

le flux d'arrivées reste continu. Construire une politique migratoire commune pérenne et résiliente est donc une nécessité. Les orientations du Conseil européen de juin, qui constituaient un compromis que beaucoup disaient impossible et qui ont été confirmées par le Conseil européen du 18 octobre dernier, sont pour nous une feuille de route qui nous engage tous. Ce plan d'action repose sur une démarche globale, couvrant l'ensemble de la chaîne migratoire, depuis les pays d'origine jusqu'à l'action sur le territoire même des États membres. Seule une démarche globale de ce type est à même de fonder une nouvelle politique migratoire, harmonisée et cohérente. Elle repose sur trois piliers : un meilleur contrôle des frontières extérieures de l'Union, le renforcement de nos règles internes et le renforcement de notre action extérieure. la réponse européenne à la crise migratoire s'appuie sur un effort significatif, réalisé ces dernières années et qui doit être amplifié, pour renforcer le contrôle des frontières extérieures de l'Union. Nous disposons aujourd'hui, pour la gestion de nos frontières extérieures, de systèmes d'information opérationnels. Le système d'information Schengen vient d'être considérablement renforcé. Le règlement sur l'interopérabilité, en discussion avec le Parlement européen, devrait faciliter la consultation des six fichiers centraux de l'Union et, partant, l'amélioration des contrôles. Le système d'entrée et de sortie devrait être opérationnel en 2020 et le système d'information et d'autorisation concernant les voyages, ETIAS, en 2021. En vue d'améliorer notre gestion commune des frontières extérieures, la Commission européenne a présenté, le 12 septembre dernier, une nouvelle proposition, que la France a accueillie favorablement, à l'instar de la majorité des États membres. de la République l'avait proposé voilà un an, de faire de l'agence FRONTEX une véritable police des frontières européenne, forte de 10 000 agents d'ici à 2020. Celle-ci serait en mesure à la fois d'apporter son soutien aux États membres subissant une forte pression migratoire et de coopérer avec les pays tiers. Le renforcement de nos moyens de gestion des frontières sera également un point important des négociations sur le futur cadre financier pluriannuel, pour lequel nous soutenons la priorité donnée à la politique migratoire dans son ensemble. la Commission plus de 30 milliards d'euros sur la période 2021-2027 pour le programme « Migrations et gestion des frontières », ce qui revient à multiplier par trois les crédits affectés à la gestion des frontières. Le deuxième pilier de la réponse européenne est le renforcement des règles internes, c'est-à-dire applicables aux migrants sur le territoire de l'Union. Comme vous le savez, la Commission a proposé au printemps 2016 une révision des sept textes constituant l'architecture du régime d'asile européen commun, dont la crise migratoire de 2015 avait mis en lumière les insuffisances. Les discussions achoppent encore sur certains points, en particulier l'équilibre entre responsabilité et solidarité, si bien que la réforme progresse de façon inégale. Deux textes sont encore en discussion au Conseil : d'une part, qui détermine l'État membre responsable du traitement d'une demande d'asile ; d'autre part, le règlement Procédures, qui porte sur les garanties procédurales pour le traitement des demandes d'asile, l'examen technique de ce dossier se poursuivant au niveau des experts. qu'un compromis soit trouvé, nous continuons à faire notre part et à participer au mécanisme temporaire mis en place cet été, qui a permis une répartition, sur une base volontaire entre États membres, des migrants ayant besoin de protection secourus en mer. Nous continuons également à travailler avec nos partenaires à Bruxelles, dans le respect du droit international et du principe de non-refoulement, à la définition des concepts de « centres contrôlés » et- je reviendrai sans le cadre des questions - non pas de « plateformes de débarquement », mais d'« arrangements de débarquement » avec les pays tiers, proposés par le Conseil européen en juin. L'approche migratoire globale inclut également le volet important des migrations légales. Nous sommes favorables à des voies de migrations sûres et légales, ainsi qu'à une politique européenne concertée à cet égard. Quant au troisième pilier sur lequel repose la réponse européenne à la crise migratoire, il s'agit du renforcement de notre action extérieure dans ce domaine. Il est essentiel de maintenir une coopération étroite et exigeante avec les pays d'origine et de transit des migrants, notamment au sud de la Méditerranée. À l'échelon régional, plusieurs forums de dialogue existent : les processus de Rabat, de Khartoum et de La Valette nous permettent d'échanger avec un certain nombre de pays africains. Ce dialogue stratégique, nous le menons aussi nous-mêmes, à l'échelle bilatérale, avec chacun des pays partenaires. plus en détail les principaux chantiers sur lesquels nous devons encore avancer avec les pays tiers. Le premier chantier est celui du renforcement capacitaire. Il s'agit de renforcer les moyens des pays d'origine pour que ceux-ci puissent mieux gérer les flux migratoires. C'est ce que nous faisons au niveau européen. Par exemple, le Maroc et la Tunisie viennent de recevoir de l'Union européenne 55 millions d'euros pour des projets de renforcement capacitaire de leurs garde-côtes ; et nous assurons nous-mêmes, à titre bilatéral, la formation des garde-côtes. Deuxième priorité : la lutte contre les trafics.

à Dakar, au Sénégal. Et nous poursuivons dans cette logique, qu'il nous faut renforcer : c'est une logique très pertinente, qui donne de très bons résultats dans la lutte contre les migrations illégales et surtout dans l'identification des passeurs. Par ailleurs,

démographique, sécuritaire, économique, voire climatique, qui sont les causes profondes des migrations. Tel est notamment l'objet du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, le FFU, doté de 4 milliards d'euros, qui a déjà permis de financer de nombreux programmes. C'est aussi dans cette perspective que le Président de la République a souhaité prendre l'initiative de l'Alliance pour le Sahel, dont

Messieurs les présidents de commission, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, contrairement à ceux qui ne cherchent qu'à entretenir cette question pour mieux l'instrumentaliser, nous agissons pour trouver, avec nos partenaires en Europe, des solutions à la fois efficaces, dignes et respectueuses des droits fondamentaux et de nos valeurs. Le phénomène des migrations est appelé à durer ; c'est en mettant en place un partenariat global fondé sur les principes que je viens d'évoquer et en incitant chaque acteur concerné à prendre ses responsabilités que nous parviendrons à maîtriser l'ensemble de cette question. Mes chers collègues, monsieur

Trois questions, monsieur le ministre. Première question, sur le paquet Asile : pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la révision du règlement Dublin ? Un débat assez ferme, si j'ai bien compris, est en cours entre l'Autriche, la France et d'autres pays sur le caractère obligatoire ou non de la solidarité et donc du partage des migrants illégaux. Je pense aussi que nous devrions avancer sur le problème du concept de « pays tiers sûr

entre l'exigence de solidarité, l'exigence de responsabilité et la nécessité de partager. Une proposition autrichienne vient d'être mise sur la table ; elle nous paraît

États tiers. Nous ne devons pas nous défausser de nos responsabilités sur les pays tiers ni créer des sortes de centres de refoulement sur la rive sud

Les urgences humanitaires ne sont toujours pas prises en charge dignement, ni en mer Méditerranée, où 15 000 migrants sont morts depuis 2014, ni aux frontières, qu'elles soient intra-européennes ou extra-européennes. Et c'est le rejet, la haine, le racisme, la répression qui continuent de progresser dans toute l'Europe. La France est-elle prête à de nouveau des initiatives importantes, non seulement sur la question sécuritaire, mais surtout sur la question de l'accueil des migrants ? Est-elle prête à sortir d'un discours qui entretient des peurs hors de proportion, prétend que la seule solution est de tenir à distance les migrants dans des centres fermés à l'extérieur de l'Union européenne ? Vous l'avez dit vous-même nous sommes passés d'un million à 115 000 entrées. Nous savons donc aujourd'hui que le pic de 2015 a déformé notre vision du problème dans la durée. Allons-nous enfin ouvrir un débat responsable

Les insécurités du monde, de toute nature, ne se régleront demain que dans l'interdépendance. Et nous avons besoin d'aborder la question des migrations sous un autre angle. Les migrations sont aussi une interpellation,

Et le texte qui va être proposé pour une meilleure gouvernance internationale des migrations est soutenu sans réserve par la France. Cette initiative émane du Mexique et de la Suisse ; nous avons accompagné ce mouvement, et nous entendons contribuer aux démarches visant à la bonne mise en oeuvre du pacte.

Monsieur le ministre, les tribunaux administratifs de Melun et de Pau ont récemment annulé le renvoi vers l'Italie de demandeurs d'asile qui avaient fait une demande en France, au regard de la politique menée par les autorités italiennes en la matière.

au dispositif des « pays tiers sûrs ». Monsieur le ministre, comment maintenir et renforcer la coopération européenne si, parmi les propositions qui circulent aujourd'hui,

M. le ministre. Monsieur le sénateur Leconte, vous évoquez la notion de « pays tiers sûr », et vous avez raison de mettre en avant la difficulté Le concept de « pays tiers sûr » se heurte, pour la France, à une double contrainte constitutionnelle : d'une part, le quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 fait obligation à notre pays d'examiner au fond les demandes d'asile des personnes se disant persécutées en raison de leur action en faveur de la liberté et, si elles relèvent de cette définition, de leur accorder une protection ; d'autre part, l'article 53-1 de la Constitution consacre le droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile à toute personne qui sollicite la protection de la France, y compris pour d'autres motifs que son action en faveur de la liberté.

l'utilisation de cette notion soit rendue facultative, afin de permettre à la France d'examiner au fond toute demande d'asile et, le cas échéant, d'accorder une protection aux « combattants pour la liberté préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par le droit national. Notre objectif, par ailleurs, est d'essayer de rapprocher autant que possible les régimes nationaux d'asile,

Leconte, pour la réplique. Monsieur le ministre, je vous remercie de ces précisions utiles. Nous partageons votre préoccupation. Toutefois, je suis très perplexe sur notre capacité

Monsieur le ministre, en m'approchant de ce micro pour aborder ces sujets difficiles que sont la sécurité, l'immigration et les frontières, j'avais en tête

Depuis le 9 mai dernier, jour où nous avons débattu de ces questions complexes devant lesquelles les opinions publiques s'irritent- je le dis avec rudesse -, bien des choses ont changé, mais nous en sommes toujours au même point. Les populismes, de l'autre côté des Alpes, en Europe centrale, en Allemagne, sans parler du Brésil, ont progressé, en six mois, à pas de géant. Même si la pression migratoire a reculé, le bras de fer entre le gouvernement italien et certaines organisations non gouvernementales a éclairé d'une cruelle lumière l'incapacité de l'Europe à parler d'une voix claire, forte et concordante sur cette question. De réunions de travail en rencontres bilatérales et en sommets européens entre chefs de gouvernement, rien n'a réellement émergé, si ce n'est que chaque État membre concerné

qu'une initiative forte de la France émerge du constat de l'échec de Dublin III, afin d'éviter que cette question ne devienne le sujet central des prochaines élections européennes

sur la nécessité d'adopter des règles internes communes ; sur le renforcement de l'action extérieure. Ces trois principes, qui engagent concrètement l'ensemble des États membres, ont été validés ; ils ont été validés

du règlement Dublin est évidemment essentielle ; il est normal qu'elle prenne un peu de temps, mais je dois constater que la présidence autrichienne, en proposant de travailler sur une solidarité

quatre ans après le début de la déferlante, nous sommes toujours en train de nous demander comment cette Europe, votre Europe, pourrait bien gérer la crise migratoire. C'est révélateur et terriblement consternant La politique, c'est d'abord la sémantique : l'utilisation du vocable « gérer », c'est-à-dire faire face, administrer démontre que votre Europe « accepte » cette déferlante permanente, et ce contre l'avis même des peuples Mais que pèse aujourd'hui la volonté des peuples face aux exigences du trafic d'êtres humains et de la finance En Marche ? C'est la lutte du pot de terre enraciné contre le pot de fric nomadisé. Car- je le dis de nouveau ici -la politique d'immigration, qu'elle soit de crise ou régulière, n'est aucunement motivée par un souci humanitaire, encore moins humaniste. L'immigration n'est qu'un outil économique : le réfugié n'est de plus en plus qu'une marchandise pour les mafias de passeurs ; l'immigré légal, quant à lui, n'est qu'un moyen, jamais une fin, au service d'un certain patronat qui trouve là le moyen d'exploiter des populations fragilisées et donc peu revendicatives pour en tirer toujours plus de profits, au détriment des peuples qui sont victimes de ce phénomène, c'est-à-dire de tous les peuples européens. L'immigration ne sert que des intérêts privés et l'idéologie chère à M. Soros, qui rêve de voir disparaître les identités nationales dans un melting-pot généralisé. Quatre ans, donc, que votre Europe est incapable de faire cesser cette crise née d'un triple chaos : chaos libyen, dont Nicolas Sarkozy est largement responsable ; chaos syrien, auquel François Hollande et Emmanuel Macron ont participé ; chaos africain, résultat de décennies de dictatures, de guerres tribales sans fin et d'une explosion démographique qui ne fait que commencer. En Italie, pays frappé de plein fouet par cette crise migratoire, l'orientation politique a changé ; elle est tournée désormais vers l'intérêt des Italiens avant tout, et les premiers résultats ne se sont pas fait attendre : les demandes d'asile y ont chuté de près de 70 % depuis que Matteo Salvini occupe le poste de ministre de l'intérieur. C'est dans cet esprit-là que mon Europe, celle du Rassemblement national et de ses alliés, agira, comme le font les gouvernements italien, autrichien, hongrois et polonais. Ma question est la suivante, monsieur le ministre : êtes-vous disposé à à quitter la table de l'idéologie pour rejoindre celle de la liberté des peuples qui, partout en Europe, clament leur volonté, et vous réclament, d'en finir avec cette folle politique d'immigration, qu'elle soit de crise ou régulière ? La parole est à M. le ministre.

y compris l'histoire italienne très récente. Ce n'est pas avec des propos de matamore qu'on réglera la question migratoire. Très bien

et l'Union européenne pour construire une gestion pérenne de l'ensemble des flux, alors nous aurons, demain ou après-demain, d'autres

est aujourd'hui mise à mal par la montée des mouvements populistes et nationalistes, qui se nourrissent du sentiment que l'Europe ne dispose plus de la maîtrise de ses frontières. La réforme nécessaire du règlement Dublin III, qui est perçu perçu comme inégalitaire par les principaux pays d'entrée, reste à ce jour sans perspective d'aboutir, en raison du blocage de certains pays. La semaine dernière, le Parlement européen a regretté que tous les efforts déployés jusqu'à présent pour mettre en place un régime de migration équitable et humain à l'échelle de l'Union aient échoué. Il a d'ailleurs décidé d'orienter une partie du budget vers la définition de solutions aux « causes profondes de la migration dans le voisinage immédiat et plus lointain de l'Union européenne ». C'est bien, n'est pas suffisant. Un tel manque de solidarité entre États, ainsi que les critiques persistantes de certains gouvernements, comme celui de l'Italie, s'inscrivent à rebours d'une démarche européenne équilibrée entre respect de nos valeurs et capacité d'édicter une règle du jeu applicable par tous.

Mais c'est la condition indispensable pour aboutir à une politique migratoire de longue durée. C'est ce à quoi nous nous employons, même s'il est un peu difficile de décliner en permanence solidarité et responsabilité. Nous avons trouvé

Monsieur le ministre, le problème des migrations à destination de l'Europe ne se joue pas que sur la Méditerranée ; d'ailleurs, lorsque les migrants ont atteint la Méditerranée, c'est qu'il est déjà bien tard tard ! La solution européenne réside aussi dans l'engagement des pays d'origine à attaquer à la racine les causes des migrations : la pauvreté, la misère, la faim, le manque de perspectives, la peur et, demain, les problèmes climatiques. L'Union européenne a pris conscience d'un tel impératif, sous l'empire de l'urgence. Elle a lancé les processus de Rabat et de Khartoum pour engager les États situés sur les routes migratoires. Elle a inclus une clause de conditionnalité dans les accords de Cotonou. En 2015, avec le sommet de La Valette, elle a établi un véritable partenariat euro-africain pour maîtriser les flux migratoires et créé le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, doté de 1,8 milliard d'euros. Vous avez évoqué ces initiatives dans votre intervention liminaire, Néanmoins, ces politiques font encore figure de rustines et d'expédients. Leur efficacité est discutable, faute d'évaluation. Et elles demeurent prisonnières d'une logique d'aide au développement, qui a démontré sa fragilité. Il convient de considérer l'Afrique comme un partenaire économique stratégique. Comme l'a dit le Président de la République à Ouagadougou en novembre 2017, il faut soutenir les entreprises africaines, créer de l'emploi, de l'activité industrielle, du commerce, et non remplir les poches d'intermédiaires ou de responsables corrompus et prédateurs.

Il y a un accord entre l'Union européenne et la Turquie, qui accueille aujourd'hui 3,6 millions de réfugiés, en provenance essentiellement du Moyen-Orient.

c'est plus compliqué à gérer qu'ailleurs. J'ai pu constater un niveau de saturation très préoccupant. Je pense qu'il faut apporter un soutien significatif aujourd'hui à la Grèce dans le cadre européen pour aider

Très récemment, plus de 200 personnes ont mené une attaque sur la frontière établie à Ceuta, qui sépare l'Espagne du Maroc. On a cru comprendre que le gouvernement espagnol voulait modifier l'organisation de cette frontière ; des déclarations ont été faites pendant l'été. En prenant

On a un peu le sentiment que l'Espagne veut gérer ou préserver ses relations bilatérales avec le Maroc et ne souhaite pas trop voir l'Europe présente dans ses discussions et sa gestion de la migration.

Le sommet européen du mois de juin 2018 s'est ainsi terminé sur une décision aussi baroque qu'incroyable pour tout humaniste : désormais, les Libyens sont responsables de la recherche et du sauvetage dans les eaux comprises entre leur pays et l'Italie ! La gestion humanitaire est donc déléguée à un pays qui ne respecte pas les droits humains ; ceux qui le fuient disent préférer « mourir en mer que vivre en Libye ». Faute de mieux, des associations ont pris le relais du sauvetage en mer depuis 2014, dont SOS Méditerranée et son navire, l'. Ils patrouillent, dans le respect du droit maritime, sur la mer devenue cimetière pour des dizaines de milliers d'êtres humains qui fuient les guerres et les persécutions. Dernièrement encore, 2 583 disparus en 2017, et déjà 1 565 morts en 2018. Cette association a permis de sauver

plusieurs milliers d'Africains qui étaient dans des camps gérés et dirigés par les passeurs, les mêmes qui allaient ensuite les envoyer en bordure de Méditerranée.

Les règles du pavillon, c'est un certain nombre de dispositions sur les équipages et la structure du bateau. Cela fait partie des règles de sécurité que nous imposons à notre propre pavillon. Pour l'instant, à ma connaissance,

! L'aide humanitaire en mer a été confiée aux Libyens, qui ne respectent pas les principes fondamentaux de l'Union européenne en matière de droits de l'homme. Et on dit à un tel pays

le traitement de la situation dans les pays d'origine, dans les pays de transfert, la gestion des frontières au sein de l'espace Schengen,

et la nécessité d'éviter les mouvements dits « secondaires ». Pourquoi y a-t-il de telles difficultés pour harmoniser le traitement du droit d'asile en Europe

est à M. le ministre. Monsieur le sénateur, l'un n'empêche pas l'autre ! Nous sommes aujourd'hui en discussion avec l'Allemagne pour que nous soyons complètement harmonisés dans nos procédures, indépendamment de l'action que nous menons ensemble pour aboutir à un résultat le plus rapide possible sur la modification du règlement de Dublin. Simplement, avec l'Allemagne,

Certes, les discours expriment une prise de conscience. Une approche globale des migrations, incluant les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne et une coopération avec les pays d'origine et de transit, ainsi qu'une nécessaire solidarité entre les États membres dans la prise en charge des flux constituent

afin de décourager les trafics et d'éviter les voyages périlleux entrepris par les clandestins. Or les activités illicites de l'- chacun comprendra ici que je ne partage pas la position de David Assouline

dont, rappelons-le, plus de 730 ont déjà péri en mer cette année. Aussi ma question porte-t-elle sur la pénalisation de ces filières clandestines hors-la-loi et sur leur éradication. Au-delà même de la politique européenne, l'article 3 du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée est entré en vigueur en 2004, c'est-à-dire il y a plus de quatorze ans. Des investigations permettent-elles aujourd'hui de connaître l'origine du financement de ces filières et de déférer les coupables à la justice ? La parole

La lutte contre les passeurs est une nécessité absolue. On n'en parle pas assez, parce que cela n'attire pas automatiquement les médias, mais c'est essentiel,

en matière de sauvetage. Dans les zones identifiées dans le cadre de cette convention, les zones de gestion disposent toutes d'un centre de coordination et de recherche opérationnelle. Il y en a un à Tripoli.

Depuis le début de cette crise, les négociations butent sur le niveau de solidarité que les uns et les autres sont prêts à mettre en oeuvre à l'égard des réfugiés entrés sur le territoire européen. Ainsi, la crise des migrants a mis en lumière les faiblesses du système d'asile européen. Pis, le poison du nationalisme se propage insidieusement dans l'Union De plus en plus, les partis hostiles à l'immigration gagnent du terrain et sèment la confusion. Cependant, le phénomène de migration n'est pas nouveau : ce qui l'est, c'est l'écho des mouvements nationaux populistes qui agitent les peurs. En Europe, ce sont « 50 nuances de brun », selon la ministre chargée des affaires européennes. Ces dernières années, la France a dû faire face à l'arrivée de plusieurs centaines de milliers de migrants. Notre pays a fait de son mieux pour donner des conditions de vie décentes à ces personnes et il faut remercier particulièrement tous les maires et les associations qui ont répondu présent à l'appel des pouvoirs publics. Je tiens à saluer l'Agence du service civique, qui a établi un programme permettant à au moins mille jeunes volontaires d'effectuer un service civique sur l'accompagnement des réfugiés, en complément de l'action des travailleurs sociaux, soit auprès d'une collectivité engagée dans l'accueil de réfugiés, soit auprès d'associations spécialisées et d'établissements publics. Il est, en effet, apparu nécessaire d'accompagner les réfugiés dès leur arrivée sur notre territoire et indispensable de les aider dans leurs démarches administratives. Monsieur le ministre, les besoins sont immenses et, afin de remplir notre mission d'accueil et de solidarité, il importe de compléter le dispositif existant, avec un système d'asile plus juste, plus simple et plus efficace : quelles solutions et quels moyens proposez-vous pour accélérer la prise en charge des dossiers des migrants ? Comment l'Europe peut-elle y participer ?

je partage votre sentiment, monsieur le sénateur : la rapidité du traitement est essentielle. C'est la raison pour laquelle les moyens de l'OFPRA ont été considérablement renforcés : l'office a vu ses moyens doubler depuis 2013

Jean-François Rapin. Monsieur le ministre, le 3 octobre dernier, Theresa May annonçait avoir présenté un projet de loi visant à mettre fin à la libre circulation des Européens au Royaume-Uni, s'engageant résolument vers une immigration choisie. immigration choisie. Qu'en est-il des migrants non européens ? À titre de rappel, Theresa May s'était engagée, dans le programme présenté pour les élections législatives de 2017, à réduire le solde migratoire à moins de 100 000 personnes par an, contre 273 000 en 2016. Cette annonce alimente la question des négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur la gestion de la crise migratoire dans le cadre du Brexit. elle fait écho à la question de la frontière territoriale entre le continent et le Royaume-Uni, qui représente un coût non négligeable pour les parties prenantes, notamment pour la région des Hauts-de-France.

nos forces de l'ordre ont de nouveau été contraintes de démanteler le camp de Grande-Synthe, afin d'enrayer les réseaux de passeurs qui organisent illégalement des traversées de migrants vers le Royaume-Uni. Je vous rappelle que, au mois de janvier dernier, Emmanuel Macron, en visite à Calais, a annoncé que les intérêts de la région seraient pleinement pris en considération dans le cadre des discussions et des négociations que la France mènera. Dans une interview accordée la semaine dernière sur la question du Brexit, Mme Loiseau déclarait que tout avait été exploré d'un point de vue technique. Néanmoins, elle ajoutait, s'agissant des consultations citoyennes sur l'Europe, que le sujet des migrations n'était pas au coeur des préoccupations des Français.

Quelle est votre position sur les accords du Touquet ? Pouvez-vous nous détailler les mesures concrètes qui sont actuellement évoquées et sur lesquelles la France se fait entendre, concernant cette gestion de la crise migratoire ? Très bien ! La parole est à M. le ministre.

Par ailleurs a été mis au point un dispositif pour accélérer les transferts vers le Royaume-Uni, en particulier pour les mineurs isolés. Enfin, un accord a été trouvé sur des actions conjointes en direction des pays d'origine et de transit, sur le modèle

qu'il faut mettre en oeuvre de manière très concrète, ont été accompagnées d'un versement britannique pour financer la sécurisation des infrastructures de transport, l'hébergement et la prise en charge des personnes vulnérables, ainsi que l'éloignement des migrants en situation irrégulière. La mise en oeuvre de ces engagements est réelle : elle progresse à un rythme qui nous paraît satisfaisant, même si l'ensemble de ces dispositifs n'a pas permis de régler l'existence de

les chefs d'État et de gouvernement ont demandé à la Commission européenne d'étudier la faisabilité de plateformes régionales de débarquement. Celles-ci prendraient la forme de financés et supervisés par l'Union européenne, et établis dans des pays tiers pour étudier la situation des migrants secourus dans les eaux internationales. dans les eaux internationales. À ce stade, les pays tiers privilégiés par les États membres pour accueillir ces plateformes, tels que la Tunisie, le Maroc et l'Albanie, ont tous catégoriquement refusé une telle coopération dans la gestion du phénomène migratoire. L'Union européenne va donc devoir engager une négociation compliquée. Il est vrai que vous êtes un spécialiste des négociations compliquées,

Les Français attendent de vous des actions concrètes pour endiguer cette immigration incontrôlée et combien préoccupante. La

qui jouent le rôle de gestionnaires potentiels de ces arrangements de débarquement, et qui ont une relation plus directe avec les autorités étatiques concernées. La parole est à M. Henri Leroy, réplique. Monsieur le ministre, si je comprends bien, vous n'irez pas plus loin avec les plateformes régionales de débarquement et vous essayerez de traiter avec chaque pays pour trouver une solution ?

je souhaiterais vous interroger sur la question des mineurs non accompagnés qui, je vous le rappelle, constitue un chantier prioritaire pour les élus départementaux, qui se sont exprimés par la voix de l'Assemblée des départements de France. En effet, l'augmentation très importante du nombre de mineurs étrangers isolés- on les appelle depuis des mineurs non accompagnés -arrivant dans nos territoires ne peut que nous interpeller. En France, le nombre de mineurs non accompagnés est passé de 5 590 en 2015 à près de 15 000 en 2017. En conséquence, les départements métropolitains font aujourd'hui part de l'état de saturation de leurs dispositifs de protection de l'enfance. À l'échelle européenne, plus de 31 000 demandeurs d'asile sollicitant une protection internationale dans les États membres de l'Union européenne étaient considérés comme des mineurs non accompagnés

Certes, la Commission européenne a affirmé que la gestion de l'asile et des migrations faisait partie de ses grandes priorités dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027, mais je regrette que la question des mineurs non accompagnés et, notamment, des « faux mineurs » non accompagnés soit traitée de façon épisodique, pour ne pas dire parfois anecdotique. monsieur le ministre, alors que nous sommes toujours en attente du plan d'action national visant à améliorer l'accueil et la prise en charge des mineurs non accompagnés et des personnes se présentant comme tels, mes questions sont les suivantes : l'Europe entend-elle

et les préoccupations des présidents de conseil départemental en matière d'accueil des mineurs non accompagnés dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Cette question prise en compte par le Gouvernement, et les ministres concernés sont tout à fait avertis et alertés de l'ampleur du problème. En réalité, on comptabilise

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de ce débat, qui a montré tout son intérêt, je crois que l'on peut retenir quelques lignes de force. Tout d'abord, les différents intervenants, que je remercie leur participation à ce débat, se sont fait l'écho des inquiétudes que ressentent nos concitoyens et, d'une manière générale, les populations du continent européen.

Comme l'ont rappelé plusieurs de nos collègues, le résultat des élections auxquelles on a assisté, notamment en Italie ou en Suède, et les événements politiques qui se déroulent sous nos yeux en Allemagne montrent bien que la question des migrations

Au-delà du droit d'asile- là aussi, les interventions l'ont bien montré -, il est ensuite absolument nécessaire de protéger nos frontières, notamment face à l'immigration économique, non pas parce que

Nous pensons véritablement qu'il s'agit de l'une des actions de fond et de l'une des priorités que nous devons poursuivre pour mettre un terme à ces migrations, faute de quoi tous les moyens coercitifs ne permettront certainement pas de maîtriser ce phénomène. Autant dire, monsieur le ministre, que nos commissions- je salue le travail qui a été fait par le président Jean Bizet et la commission

des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d'être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de l'exercice de leur métier ou de leurs fonctions. fonctions. Débat sur le préjudice représenté, pour les entreprises françaises, par la surtransposition du droit européen en droit interne. Débat sur le financement de l'accompagnement médico-social des personnes handicapées. Personne ne